dans les établissements scolaires en ce début d'année, en raison du variant omicron, qui fait bondir le nombre de contaminations à un niveau encore jamais atteint. Les cas positifs se multiplient dans les écoles et le nombre de fermetures de classes commence à augmenter. Or il nous paraît absolument impératif de limiter au maximum la circulation du virus en milieu scolaire. Cet amendement tend à donner au Premier ministre la faculté d'instaurer une politique de dépistage régulière, avec des campagnes de tests salivaires dans les écoles et la distribution d'autotests pour les collégiens.

destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d'activités, quant à la stratégie vaccinale à mettre en oeuvre pour limiter la quatrième vague de la pandémie, rapport que notre collègue Bernard Jomier a déposé le 1 juillet dernier.

et très difficile, madame la présidente, pour les parents comme pour les enseignants. C'est pourquoi vous comprendrez l'importance de cet amendement ! Il s'agit donc de l'amendement

le régime de gestion de la crise sanitaire permet déjà de faire ce que vous proposez. Je ne tiens pas à ce que nous rigidifions davantage encore un système qui a fait la preuve de sa complexité. D'ailleurs, cette

que la communauté nationale prenne en charge une campagne de dépistage dans les écoles élémentaires

dans la recherche d'un compromis moins néfaste pour la sauvegarde de nos libertés publiques dans un temps de crise sanitaire qui plonge notre pays dans un état d'exception depuis près de deux ans.

virus ? On peut certes espérer, avec les plus optimistes, que le variant omicron sera le dernier, mais c'est loin d'être certain. Bref, tout cela est hypothétique et vous le savez sans doute mieux que nous. L'effort dialectique est donc considérable, mais il ne nous convainc absolument pas.

Noël. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'alinéa 6 conditionne l'accès à certains établissements à la détention d'un justificatif de statut vaccinal, malgré les nombreuses promesses du Gouvernement de ne jamais recourir à un tel dispositif. Cette exclusion assumée des citoyens non vaccinés est inacceptable. En instaurant un passe vaccinal, le Gouvernement entrave les libertés les plus fondamentales en se dotant d'un outil de discipline à l'égard de n'importe quel citoyen, en fonction de son statut vaccinal. Le passe vaccinal s'appuie sur une triple hypocrisie. Premièrement, dans la mesure où la vaccination n'est pas obligatoire, le choix d'une partie de nos concitoyens de ne pas y recourir ne saurait emporter une quelconque forme de déchéance de citoyenneté. On ne peut pas les sanctionner pour un choix qui ne constitue pas un délit. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres, le « en même temps » vaccinal est un échec et une escroquerie ; il se traduit par la négation de toutes les valeurs de notre République. Deuxièmement- faut-il le rappeler ? -, plus on a besoin du vaccin, moins on a besoin du passe vaccinal. Nous avons maintenant une connaissance plus fine de ce virus et nous savons que ce sont les sujets âgés ou atteints de comorbidités qui développent les formes les plus graves. La mortalité, faible en dessous de 50 ans, augmente progressivement chez les sujets âgés de plus de 65 ans, qui représentent plus de 80 % des décès. Croyez-vous vraiment que la mise en oeuvre d'un quelconque passe vaccinal à l'entrée des discothèques, des parcs d'attractions, des piscines, des bibliothèques ou des bars poussera ces sujets fragiles à la vaccination ? Absolument pas

Le Gouvernement partage la volonté du Sénat d'encadrer de la manière la plus équilibrée possible la mise en oeuvre de ces outils nécessaires à la lutte contre l'épidémie ; les évolutions du projet de loi

vaccinal est la solution la plus à même de nous prémunir de restrictions plus importantes encore des libertés. Pour ces raisons, le Gouvernement estime que l'encadrement du recours à ce dispositif est poussé à son maximum dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, à laquelle je vous propose donc, par cet amendement, de revenir. Pour les mêmes raisons, le recours au passe sanitaire, et non pas vaccinal, pour la tenue de réunions politiques, ne peut être conditionné à de tels critères stricts et rigides, qui ne permettent pas une adaptation rapide des moyens de lutte contre l'épidémie.

méritent une attention particulière, et je suis bien placé pour défendre ce point de vue. Il est en effet nécessaire de garantir leur accès à des activités indispensables à leur développement, comme les sorties scolaires ou les activités périscolaires

Ce que nous propose notre rapporteur, et qui a été soutenu par la commission, consiste à créer un automatisme de disparition de la réglementation du passe vaccinal, en fonction du franchissement de certains chiffres d'évolution de la pandémie.

Comment sera-t-il vérifié ? Quelle est la date de l'obligation d'abrogation du décret ? Qui en a la responsabilité ? Rien de cela n'est prévu. Le système est en outre anormalement rigide, puisque,

Ce n'est évidemment pas du tout fonctionnel. Enfin, cette rédaction crée une mosaïque totalement irréaliste en entendant appliquer le décret

l'on change de chiffre. Tous les éléments de la vie quotidienne de nos compatriotes, qui les conduisent à se déplacer d'un département à un autre, en seraient évidemment perturbés. Il me semble que cela a été conçu de manière trop artificielle, avec l'objectif politique de manifester une différence avec le Gouvernement. Il vaut beaucoup mieux conserver la méthode réaliste que le rapporteur a défendue, par exemple, à propos de la capacité des stades,

L'article 1 du présent projet de loi vise à transformer le passe sanitaire en passe vaccinal, plus restrictif. Lors des débats en commission des lois, un amendement du rapporteur a permis de définir des critères d'extinction de ce dispositif.

au fait que l'hôpital ne doit pas voir la pression s'accentuer sur lui avant d'avoir repris un mode de fonctionnement normal, c'est-à-dire

trois critères : le nombre d'hospitalisations au plan national, la vitesse de circulation du virus au plan local, mais aussi le nombre de personnes vaccinées au plan local. Quand beaucoup de gens sont vaccinés et que le virus circule peu, si l'hôpital n'est pas sous une tension excessive au plan national,

et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. » Il me semble que, en bonne législation, cette formulation est suffisante ; elle remet la responsabilité entre les mains du Gouvernement, sous le contrôle du juge

s'il n'a pas de conséquence sur le système de santé, sur les hôpitaux, s'il ne conduit pas à des déprogrammations, s'il n'entraîne pas 30 000 hospitalisations, il

Je voudrais dire à notre collègue Alain Richard que je partage naturellement sa confiance à l'égard du juge. Pourtant, entre un contrôle exercé par le juge et un contrôle exercé par le Parlement, lequel limite les pouvoirs

d'État : votre gouvernement a abandonné volontairement la bataille contre la propagation du virus, dont les conséquences seraient atténuées par un vaccin protecteur évitant les formes graves, en misant tout sur une circulation de plus en plus importante

puisqu'il s'agit de chiffrer, non pas le nombre de malades, mais le nombre de cas. En effet, pour rendre compte de la situation épidémique réelle, un test positif doit être corrélé à des signes cliniques.

Introduire le suivi des cas symptomatique en s'appuyant sur les réseaux classiques de suivi des épidémies permettra de contrôler de manière plus pertinente la réalité de la situation épidémique sur le territoire.

publics doivent être mises en oeuvre dans une perspective de réduction des inégalités sociales et territoriales.

appliquée de manière à réduire les inégalités territoriales et sociales. Croyez bien, cher collègue, que la commission fait sien l'objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales dans l'accès à la vaccination. Toutefois, il ne me semble pas qu'on qu'on puisse placer cet objectif au même niveau que les objectifs de rétablissement de la sécurité sanitaire face à la propagation de l'épidémie, qui relèvent de pouvoirs exceptionnels. L'avis est donc défavorable.

sensibilisation des médecins traitants pour les inciter à proposer la vaccination à domicile, mise en oeuvre d'opérations de vaccination dans les centres d'hébergement d'urgence, dans les hôtels sociaux et dans certaines universités, organisation de permanences dans des relais alimentaires associatifs pour aider à la prise de rendez-vous, prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport vers un cabinet médical ou un centre de vaccination pour les personnes qui rencontrent des difficultés à se déplacer. Au total, monsieur le sénateur, Au total, monsieur le sénateur, lors du bilan qui a été réalisé le 7 octobre dernier, il y a donc plus de trois mois, on dénombrait déjà plus de 4 000 opérations de ce type ciblées sur les personnes précaires et sur les personnes éloignées de notre système de soins et de vaccination.

Par souci d'égalité, il est proposé d'appliquer aux étrangers souhaitant résider dans notre pays pour une durée d'au moins trois mois les mêmes restrictions que celles qui pèsent sur les Français. En effet, il ne faudrait pas que les Français soient les plus mal lotis chez eux. Cette précision de bon sens entraîne une conséquence évidente : en cas de non-respect de cette obligation, les étrangers feront l'objet d'une décision administrative d'obligation de quitter le territoire français, telle que la définit l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

car ils ne sont déjà plus des citoyens -non plus de seconde zone, mais de troisième zone dans leur propre pays. J'en appelle donc à la cohérence et à l'égalité de tous : nous sommes tous égaux devant la loi, y compris devant la loi de l'emmerdement maximal.

Cette précision est nécessaire, car la vaccination contre la covid-19 a été proposée en priorité aux groupes vulnérables, puis étendue à plusieurs catégories de la population. Pour toute personne souhaitant se faire vacciner, il faut s'assurer qu'elle soit éligible, c'est-à-dire qu'elle fasse partie des groupes prioritaires et qu'elle ne présente pas de critères d'exclusion. ne présente pas de critères d'exclusion. Avec le temps, les groupes prioritaires ont évolué en fonction de l'avancée de la campagne de vaccination. En outre, les critères d'exclusion sont également susceptibles d'évoluer en fonction des types de vaccins disponibles et de l'avancée des connaissances médicales.

les paramètres de la prise en compte du nombre de vaccinés pour la décision d'appliquer ou de ne pas appliquer le passe vaccinal.

Christian Klinger. L'article 1 du présent projet de loi vise à transformer le passe sanitaire en passe vaccinal, ce dernier étant plus restrictif que le premier. il est regrettable que le dépistage virologique et le certificat de rétablissement soient désormais totalement exclus au profit du seul statut vaccinal. Cette Cette mesure n'aura d'autre effet que de resserrer l'étau liberticide que le Gouvernement resserre un peu plus à chaque texte d'urgence sur la crise sanitaire. En conséquence, il est nécessaire d'en circonscrire au maximum l'utilisation et d'en définir les modalités d'application. En passant du passe sanitaire au passe vaccinal, le Gouvernement fait le choix de se passer des tests, alors que c'est un outil plus fiable pour garantir la non-contagiosité. Le présent amendement vise donc à laisser aux Français les plus jeunes, et donc les moins à risque, la liberté d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas malades par un autre moyen que le seul statut vaccinal. Par cet amendement, nous proposons de réserver l'application du passe vaccinal aux seules personnes de plus de 50 ans. que nous avons retenu correspond à l'âge à partir duquel on observe une nette augmentation du taux d'hospitalisations en soins critiques ces dernières semaines.

l'inefficacité du vaccin sur la propagation du virus a été prouvée par l'observation scientifique. De nouveaux records de contaminations ont été atteints dans notre pays, alors même que la grande majorité des Français est vaccinée.

tandis que les 0-19 ans représentent 0,02 % des décès hospitaliers et 0,6 % des personnes admises en réanimation. Les moins de 40 ans ne sont donc pas le public le plus touché par les dangers de cette maladie. De plus, le 8 novembre 2021, la Haute Autorité de santé déconseillait aux personnes de moins de 30 ans de se faire administrer le vaccin du laboratoire Moderna.

atténuer le risque d'exposer les professionnels à des tensions avec leurs clients et réduire leur charge de travail, en intégrant dans le dispositif du passe sanitaire une photographie de son titulaire.

vaccinal. Cette solution moins attentatoire aux libertés individuelles et plus opérationnelle permettrait de supprimer dans le présent texte les alinéas prévoyant le contrôle d'identité par les personnes chargées de vérifier le passe vaccinal.

Imposer la photographie du titulaire sur le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 permet de limiter les risques d'usurpation d'identité et d'usage frauduleux de ce document, garantissant ainsi une meilleure prise en charge, le cas échéant. En outre, ce document alliant photographie, nom et prénom de la personne renforce la transparence et permet de protéger l'ensemble des personnes présentes dans les lieux soumis au passe vaccinal en garantissant, à l'instant , la situation vaccinale et sanitaire de chacun.

conformément aux préconisations du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), dont le président, Jean-François Delfraissy, déclarait : « Le passe sanitaire ne doit pas concerner les adolescents et les enfants. [ ...] Le recul existant ne permet pas d'assurer la pleine sécurité de ces nouveaux vaccins chez l'adolescent. » Les conséquences de la pandémie sur la santé psychologique et mentale des enfants, et surtout des adolescents, sont profondes et probablement durables. » Il concluait ainsi : « S'agissant de l'immunité collective, est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes de bénéfice collectif, du refus de la vaccination d'une partie de la population adulte ? Le bénéfice des vaccins pour les enfants et les adolescents n'est pas avéré, les adolescents développant moins de formes graves. En France, les moins de 18 ans représentent 1,1 % du total des hospitalisations et 0,9 % du total du total des admissions en soins critiques. Le recours aux vaccins pour la tranche 12-18 ans était initialement préconisé pour empêcher la transmission du virus au reste de la population. Ce n'est plus justifié, puisque le vaccin n'empêche pas cette transmission. Le rapport bénéfice-risque de la vaccination chez les plus jeunes n'étant pas démontré, il convient de faire preuve de la plus grande prudence et de ne pas inciter inutilement à les faire vacciner.

Si elle retire à des personnes le droit de pouvoir se déplacer, d'exercer des activités, alors même qu'elles ne peuvent pas se faire vacciner, la loi sera à l'origine de traitements inéquitables au sein de la population française. Le législateur doit donc prévoir des outils de substitution pour des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison de troubles ou de pathologies qui seraient incompatibles avec la vaccination contre la covid-19.

Résultat : ces personnes attendent très longtemps pour faire un test d'allergie et voir si elles peuvent ou non se faire vacciner. Pour éviter cette situation, une attestation personnelle délivrée par l'ARS dont elles dépendent, sur prescription du médecin traitant, devrait leur accorder une dérogation pour leur permettre de continuer d'exercer leurs activités et d'entrer dans les lieux recevant du public grâce à un test virologique de moins de soixante-douze heures ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Tel est l'objet de cet amendement. L'amendement

de la mesure pour limiter la propagation de l'épidémie. Il a estimé que le contexte sanitaire, en particulier la diffusion du variant omicron, pouvait justifier ce renforcement des mesures de protection dans les transports de longue distance.

de maintenir la solution du passe sanitaire, qui est déjà en vigueur. Vous le savez, le projet de loi impose le passe vaccinal pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, avec une dérogation prévue uniquement en cas de justification d'un motif impérieux d'ordre familial, de santé, depuis les travaux de notre commission des lois, d'ordre professionnel. Dans ce cas, la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sera demandée. En cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis, ces dispositions ne s'appliqueront pas. La présente disposition, nous semble-t-il, soulève de sérieuses difficultés : que faut-il entendre par motif impérieux ? Quels seront les justificatifs susceptibles d'être admis par les responsables chargés de contrôler les documents ? Comment les contrôleurs et les contrôleuses vont-ils apprécier ces motifs ? L'imposition du passe vaccinal pour l'accès aux services de transport visés par le projet de loi porte, à notre sens, directement atteinte à la liberté d'aller et venir et, potentiellement, par ricochet, à d'autres droits, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale. Or de telles restrictions doivent s'avérer non seulement nécessaires, mais également proportionnées. Il s'agit de prévoir des mesures qui concilient au mieux l'objectif visé, à savoir la protection de la santé publique, et l'exercice des droits et libertés. Certes, le brassage de populations qu'entraîne un parcours de longue distance constitue un facteur de risque de diffusion du virus. Pour autant, ce n'est pas un fait nouveau et aggravant justifiant l'adoption d'une mesure plus restrictive. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a expliqué le ministre de la santé à l'Assemblée nationale, les personnes ne disposant pas d'un passe vaccinal ne pourront pas forcément utiliser un autre moyen de transport. Aussi, pour que l'ensemble des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas vaccinés, mais qui présentent un test négatif, puissent circuler, il faut adopter cet amendement.

Dans ce cas précis, la restriction de liberté est manifestement disproportionnée par rapport au but de protection de la santé. Permettez-moi de parler de mon propre cas de citoyen et de parlementaire, vous invitant de la sorte à mesurer l'inconstitutionnalité de cette mesure. En dehors du fait que je suis membre du Rassemblement national, que je bois du café debout au bistrot, que je mange et bois dans le train, comme mon métabolisme me l'impose, je ne suis pas vacciné. Je sais, je cumule beaucoup de tares et de flétrissures, mais c'est ainsi Je devrai donc, dès la semaine prochaine, prendre ma voiture pour faire huit heures de trajet aller et huit heures de trajet retour pour examiner la loi, voter et contrôler l'action du Gouvernement. Avouez, mes chers collègues, que le bilan carbone, sachant qu'en plus

Je suis donc matériellement dans l'incapacité de remplir mon rôle de législateur. Faut-il en conclure que vous êtes en train de voter une obligation vaccinale déguisée non assumée Pas le droit de monter dans le train, parce qu'on n'est pas vacciné. Pas le droit de prendre la voiture, car ce serait se rendre coupable d'un écocide. Pas le droit de venir au Sénat à cheval, une atteinte au droit de l'animal. Ce monde que vous nous offrez devient fou ! Vous ouvrez une boîte de Pandore. On va tous finir à pied, mais jamais en marche mandat parlementaire exercée à mon encontre par ce texte ne saurait cacher la situation de très nombreux Français, travailleurs et familles, non vaccinés, c'est-à-dire n'ayant reçu aucune,

de dispenser d'un passe sanitaire les personnes effectuant des déplacements interrégionaux pour des motifs impérieux, familiaux ou de santé. Ni justificatif de vaccination ni test négatif n'était alors demandé. Nous souhaitons donc que cette mesure soit conservée.

est à Mme Sylvie Robert. Le présent amendement vise à maintenir la possibilité de présenter un test négatif pour les personnes en situation d'apprentissage, lorsqu'elles doivent se déplacer par transports interrégionaux dans le cadre de leur formation. compléter l'exclusion des personnes auxquelles l'activité professionnelle ou la recherche d'emploi impose des déplacements de longue distance du champ de l'application du passe vaccinal, exigé comme unique justificatif. L'absence de dérogation à cette restriction pourrait aboutir à une discrimination des apprentis fondée sur leur lieu de résidence. En effet, un employeur pourrait souhaiter éviter de signer une convention avec un apprenti

pour se rendre dans un établissement de santé, social et médico-social, pour des soins programmés. Cette obligation concerne les malades comme leurs accompagnants. Alors que, en l'absence de lits et de personnels formés supplémentaires depuis deux ans, les hôpitaux sont contraints de déprogrammer les interventions et retardent les prises en charge des patients, l'obligation de présenter un passe sanitaire aggrave le phénomène de renoncement aux soins et les conséquences des pathologies. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition. : La parole est à Mme Sylviane Noël. Les mesures restreignant l'accès aux services et aux établissements de santé contreviennent aux principes fondamentaux de la Constitution. L'accès aux soins doit être libre et garanti pour l'ensemble des citoyens du territoire. De surcroît, l'application du passe sanitaire pour accéder aux soins est un non-sens d'un point de vue sanitaire. Il restreint la possibilité pour les citoyens de se faire soigner et des dérives ont été constatées ces derniers mois. Le vaccin ne permettant pas de garantir une non-contagiosité des patients ou visiteurs à l'hôpital, la mesure ne paraît pas justifiée. Je rappelle encore une fois que l'application du passe sanitaire coûte chaque mois 60 millions d'euros

est à Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement de repli vise à exclure les consultations en santé mentale, les soins psychiatriques, psychologiques et psychothérapeutiques de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire. Alors que la pandémie a fortement détérioré la santé mentale de nos concitoyennes et de nos concitoyens, il semble indispensable de maintenir l'accès aux professionnels de santé mentale.

de passages à l'acte auto-agressifs, qu'il s'agisse de tentatives de suicide, de scarifications, d'automutilations, de conduites à risque. Ce sont des signes de détresse et de désespoir liés à des tendances anxieuses anxieuses et dépressives. Les consultations en centre médico-psychologique ou directement en établissement psychiatrique doivent demeurer ouvertes sans obligation de présentation d'un passe sanitaire. Il s'agit d'un impératif de santé publique,

et au passe vaccinal pour les autres activités de loisir. C'est une usine à gaz, un dispositif confus, voire hypocrite, lorsque l'on sait que de nombreuses sorties et activités scolaires ont été annulées en raison du regain de l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui. Par ailleurs, la justification sanitaire de ces dispositions n'a pas été clairement établie, comme le souligne le rapport de la commission de lois, qui a supprimé l'obligation de passe vaccinal pour les mineurs. Cependant, nous souhaitons aller plus loin et exclure clairement les mineurs de moins de 18 ans de toute obligation de présentation d'un passe vaccinal ou sanitaire. L'amendement n° 125 rectifié,

à la covid-19 sans cumuler ce critère avec la notion de schéma vaccinal complet ou de circulation active du virus. En effet, une circulation active ou une faible couverture vaccinale n'entraîne pas une hausse des hospitalisations proportionnelle. C'est le cas aujourd'hui avec le variant omicron, qui a infecté un très grand nombre d'individus- on dénombre autour de 300 000 contaminations par jour -, y compris des personnes disposant d'un schéma vaccinal complet. Fort heureusement, il se révèle moins dangereux que d'autres variants.

Cette disposition nous paraît tout à fait déséquilibrée. Les bibliothèques et les médiathèques sont des lieux d'échange et de lien social. Ces lieux concourent à l'apprentissage et à l'éducation de nos enfants et adolescents. Si les gestes barrières sont respectés dans ces établissements, il n'est nullement besoin d'en subordonner l'accès à la présentation d'un à la présentation d'un passe, tant vaccinal que sanitaire, pour les jeunes de moins de 18 ans. Cette proposition vise donc à protéger l'ensemble des enfants et des adolescents, qui subissent de plein fouet les conséquences économiques et sociales de la pandémie de covid-19. : La parole est à M. Patrick Chaize. L'article 1 du projet de loi introduit la possibilité pour le personnel ou le responsable du lieu, de l'événement ou de l'établissement, de « contrôler l'identité » du titulaire du passe, en cas de doute, par la production d'un document officiel d'identité. Ce « contrôle d'identité » risque de mettre le gérant d'un établissement ou d'un événement en situation délicate, dès lors qu'il ne dispose pas de motifs impérieux réels ou d'une délégation de police pour contrôler l'identité d'un client ou d'un visiteur. La photo du titulaire du passe, répondant aux normes de production biométriques, permettrait de garantir l'authenticité de l'attestation, tout en facilitant la gestion des flux et des entrées pour les exploitants. Une photo réalisée en comportant de vrais risques de fraude, celle-ci devrait plutôt répondre aux normes biométriques ISO et être réalisée dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

à un décret simple n'est pas acceptable. En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition. Par cet amendement, nous souhaitons alerter nos collègues sur les nombreux renvois au pouvoir réglementaire de mesures complémentaires au passe vaccinal contraignantes pour la population et restreignant l'exercice des libertés. Tel est le cas de la détermination des situations qui exigeraient la présentation d'un passe vaccinal renforcé, figurant à l'alinéa 19 de l'article 1 du présent texte. Ce mécanisme s'inspire de ce qui existe en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Suisse, et il risque de s'appliquer prochainement, le Gouvernement envisageant de le mettre

Il nous apparaît disproportionné de décider par voie réglementaire d'une restriction supplémentaire pour l'accès à certains lieux. Ce « passe + » nous paraît incongru dans ce texte. Nous vivons aujourd'hui des records de contamination sans que le Gouvernement ait jugé nécessaire de prendre, dès début décembre, des mesures de freinage, comme le préconisait le conseil scientifique.

Nous refusons de lâcher la bride au Gouvernement pour décider seul de telles restrictions, dont la proportionnalité reste encore à démontrer.

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'exiger la présentation cumulée d'un justificatif de statut vaccinal et d'un test négatif. Cette mesure est en effet prévue à l'article 1 de ce projet de loi, qui confie le soin à un décret de définir le champ d'application des activités relevant de cette double présentation. Le Gouvernement envisage ainsi de se réserver, sans contrôle du Parlement, la possibilité d'exiger un cumul de justificatifs lorsque l'intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire l'exigent, un cas de figure qui laisse une très grande marge d'appréciation à l'exécutif. Nous aurions préféré que ces circonstances soient précisément énoncées dans ce projet de loi. M. Véran a cité le cas des discothèques lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, mais que savons-nous du champ d'application qui sera,, ainsi défini ? Nous refusons cet excès de pouvoir réglementaire et souhaitons supprimer cette disposition, qui, à notre sens, prive le Parlement de ses pouvoirs. Par ailleurs, si vous voulez, comme vous l'affirmez, favoriser la vaccination, il faut effectivement lui donner du crédit et du sens. Nous pensons pour notre part que cette vaccination a effectivement tout son sens, mais il convient de démontrer à celles et à ceux qui ont fait le parcours vaccinal, comme vous le souhaitez,

présenté comme la solution miracle à la crise sanitaire par le Gouvernement, ce dernier vient d'introduire la possibilité de mettre en place, par décret, des mesures restrictives Ainsi, en fonction de l'appréciation de la situation sanitaire, l'exécutif pourra exiger par décret, en plus de la présentation d'un schéma vaccinal complet, la présentation de résultats de tests de dépistage négatifs pour accéder à certains lieux. Dans le dernier avis relatif à ce projet de loi, la Défenseure des droits se dit particulièrement inquiète du renvoi au pouvoir réglementaire pour l'adoption de mesures complémentaires contraignantes pour la population. Elle ajoute, à juste qu'il appartient au seul législateur d'adopter ces mesures et de les encadrer. J'estime qu'il est indispensable pour la représentation nationale de débattre afin de déterminer si davantage de mesures contraignantes doivent être envisagées en cas de dégradation de la situation.

pour revoir en profondeur la stratégie autoritaire et contraignante que développe le Gouvernement depuis près de deux ans. Je demande donc la suppression de cet alinéa.

tant pour les exploitants, qui n'auraient plus à exiger de leurs clients la présentation d'un deuxième document, que pour les clients eux-mêmes, qui verraient cette opération simplifiée. Cette proposition revient donc à introduire une simplification pour tous dans la mise en oeuvre des passes sanitaire et vaccinal.

concordance documentaire en cas de doute sur l'authenticité du document. Rappelons que l'inclusion d'une photographie d'identité a été légitimement réclamée par les acteurs du secteur de la restauration et de l'hôtellerie pour faciliter leur mission de contrôle. Les

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la vérification d'identité lors de la présentation du futur passe vaccinal. Si la fraude sur ces documents doit être sévèrement combattue et punie, ces dispositions viennent renforcer le sentiment d'une défiance du Gouvernement à l'égard des Français.

Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur ne justifie pas d'étendre cette vérification. Pour ces deux motifs, il convient de laisser cette tâche aux autorités dont c'est le métier : les forces de l'ordre.

le principe d'un contrôle d'identité réalisé par des personnes non habilitées à le faire. Qui plus est, ces personnes ne souhaitent pas effectuer ces contrôles ! En outre, on leur laisserait une pleine appréciation, à leur discrétion totale, des critères selon lesquels ils pourraient ou non contrôler ces papiers.

ces contrôles. Or la viabilité du passe vaccinal dépend grandement de son contrôle. Le texte adopté par l'Assemblée nationale permettait d'octroyer aux personnes chargées de ce contrôle le droit d'effectuer non pas un contrôle d'identité, mais une « vérification de la concordance entre Si cette astuce lexicale n'a pas été conservée par la commission des lois du Sénat, le dispositif adopté par celle-ci reste tout de même problématique. La rédaction retenue laisse toujours aux personnes aux personnes chargées du contrôle du passe vaccinal la possibilité d'effectuer un contrôle d'identité. Ce transfert de compétence de la police vers la société civile n'est pas acceptable. Comment se prémunir de possibles discriminations ? Comment éviter les abus, volontaires ou non, de la part de ceux qui devront effectuer ces contrôles ? Une grande majorité d'entre eux ne sont ni formés ni qualifiés pour ce faire. Ajoutons à cela l'aspect chronophage d'un tel contrôle, plus lourd que le scan d'un QR code, qui peut le rendre difficile à réaliser dans certains établissements. Cette question du contrôle de l'identité ne semble être

être adoptées, nous permettrions à chacune et chacun, en l'espace d'une nuit, de devenir officier de police judiciaire et de contrôler tout le monde

dans les lieux dont l'accès est assujetti à la présentation du passe sanitaire une vérification allégée de la correspondance entre le passe sanitaire et

quand un doute évident apparaissait au responsable de l'accueil dans ces établissements. En outre, il convenait d'y mettre une condition importante, à

le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel à prévoir que les exploitants d'établissements recevant du public puissent exiger la présentation d'un document officiel.

qui se trouvent dans les établissements de santé et dont l'état nécessite une prise en charge sanitaire ou médico-sociale. Ces personnes présentent des risques importants de contracter une forme grave de la maladie, ce qui justifie la mise en oeuvre de protections à l'égard du virus. Je rappelle également que cette obligation n'est applicable qu'aux personnes qui accompagnent les personnes accueillies dans ces services de santé et les personnes accueillies pour des soins programmés ou qui leur rendent visite. Elle ne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

qui visent à supprimer la possibilité pour les exploitants d'établissements de procéder à une vérification de concordance entre l'identité du détenteur d'un passe vaccinal ou sanitaire et les données nominatives figurant sur un